L'ordre du jour appelle les réponses à des questions orales. La parole est à monsieur Pierre-Antoine Levi. Je vous en prie, chers collègues. Merci monsieur le président, mes chers collègues, monsieur le Ministre. L'État a fixé comme objectif de réduire de 40% la consommation d'énergie des bâtiments publics chantier évalué à près de 40 milliards d'euros. Les collectivités locales souscrivent bien évidemment à cet objectif. Pour des raisons écologiques. Tout d'abord car tout le monde a pris conscience de l'urgence climatique. Les dernières années nous l'ont suffisamment démontré. Mais la raison est également financière car des bâtiments rénovés thermiquement sont synonymes de belles économies dans un contexte où la facture énergétique pèse très lourd dans le budget des communes. Dans ce bâti en besoin de rénovation thermique, les écoles, les collèges et les lycées sont souvent en haut de la liste des collectivités le souhaitent mais beaucoup ne le peuvent pas. Dans de trop nombreux établissements les élèves doivent s'emmitoufler l'hiver et garder leurs manteaux était par contre certaines classes sont de véritables étuve. Cette situation n'est pas acceptable dans notre pays en 2023. Pour remédier à cette situation difficile pour la jeunesse, les collectivités ont besoin d'un soutien car beaucoup ne peuvent pas supporter à elle seule le coût des travaux. L'État contribue certes au travers de la décile et de l'adultère. Mais il arrive souvent que les 20 à 30% restants à financier demeure insupportables pour les Budgets communaux. Par ailleurs, compte tenu de la forte hausse des matières premières. Il arrive régulièrement que les collectivités doivent renoncer à leur projet étant souvent incapables d'auto-financiers, la forte augmentation. J'ai interrogé il y a quelques semaines, la ministre des collectivités territoriales à ce sujet. Monsieur le Ministre, comment comptez-vous faire pour appuyer de façon encore plus importante. Les collectivités dans leur démarche de rénovation énergétique, notamment des bâtiments scolaires. Ce serait un vrai signal que vous donneriez à l'ensemble des maires. La transition écologique ne doit pas être réservé aux seules communes les plus aisés. Je vous remercie. Merci. Collègue, la parole est à monsieur Clément Beaune. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Lévy vous interroger le gouvernement sur ce sujet en effet essentiel est difficile dans le contexte actuel sur les coûts de l'énergie sur la rénovation énergétique des bâtiments publics et en particulier du bâti scolaire et la situation des plus petites collectivités, vous avez raison, doit à cet égard faire l'objet d'une plus grande attention encore l'État apporte un soutien déjà important au projet de rénovation thermique des bâtiments des collectivités. Vous l'avez dit brièvement, ces projets sont d'abord éligibles à la décile et à la DETR qui sont maintenus à un niveau extrêmement élevé même historiquement élevé en 2023. Les bâtiments ont bénéficié aussi du plan de relance, avec la décide décide décide dites rénovation thermique dans les compartiments spécifique dont le montant a atteint près d'un milliard d'euros, 950 millions pour être précis. En 2021, ainsi que à travers une déciles exceptionnelle qui a aussi permis d'apporter un soutien complémentaire de 950 millions d'euros, là encore les collectivités qui bénéficient de ces différents soutiens de l'État doivent participer cofinancé dans ces transformations ces rénovation à hauteur de 20%, avec toutefois un certain nombre d'exceptions prévues pour certains investissements pour justement de tenir compte de circonstances exceptionnelles, ou de nature spécifique et coûteuse de certains projets. C'est notamment le cas des monuments protégés dont on sait qu'il s'agit souvent l'opération sensible complexe complexe pardon et onéreuse. J'ajoute que ses soutiens sont complétées par les attributions de FCTVA. Qui sont susceptibles d'être versés pour les dépenses éligibles, ce qui là aussi vient diminuer le reste à charge pour des collectivités notamment des petites communes en 2023 à travers le Fonds Vert que porte le ministre Béchu nous pourrons rehaussé en fonction des projets ses soutiens. Mais on doit réfléchir aux modalités de financement de ces travaux de manière plus générale, vous avez raison c'est notamment l'objet de la proposition de loi adoptée à l'Assemblée nationale sur le tiers-financement qui a été discuté cette semaine au Sénat sur la rénovation thermique car qu'on rénove les écoles c'est à la fois une nécessité un soutien indispensable aux communes que nous renforcerons et puis un cercle vertueux ou les dépenses d'investissements d'aujourd'hui font des économies de fonctionnement de demain également. Merci, monsieur le Ministre, Monsieur Lévy un droit de réponse. Oui, rapidement. Merci pour votre réponse Monsieur le Ministre, moi je souhaite réellement vous alerter sur la volonté des maires, surtout des petites communes de Rhino de rénover leurs bâtiments scolaires, mais elle ne peut vraiment pas le le faire compte tenu des hausses des matières premières, ne peut-on pas imaginer portée de 80 à 90%. Exceptionnellement, le montant des des cofinancements. Merci monsieur Lévy. La parole est à madame Martine Berthet. Merci monsieur le président. Monsieur le Ministre, chers collègues, je souhaite attirer Monsieur le Ministre votre attention sur les enjeux et les conséquences du projet de zone spéciale de carrières de gypse d'anhydride dans la vallée de la Maurienne. Si je conçois l'importance des enjeux de ce projet qui permettrait de gagner en autonomie grâce à un approvisionnement durable en matières premières. Je m'interroge sur l'ampleur de la zone retenue pour 120 ans et sur ses impacts sociaux, environnementaux et économiques en effet le périmètre prévisions prévisionnel pardon de la AZ. Recoupe 404 hectares dans la vallée de l'Arve en 627 en Haute-Maurienne dont une grande partie autour du village de vraiment qui se retrouvent complètement englobé. Cette zone est extrêmement large, quand on connaît le territoire très contraint qui est celui de la Maurienne. Celle-ci accueille déjà plusieurs carrières. Elle est très sollicité par le chantier de la liaison ferroviaire européenne Lyon Turin et participent ainsi déjà largement à l'effort national. Il n'est pas envisageable pour ses habitants et ses élus que leurs valises soient sacrifiés. La la vallée de la Maurienne dispose d'un Patrimoine naturel paysagé historique culturel exceptionnel et très riche, permettant à de nombreuses activités agricoles et touristiques de prospérer, comme par exemple la station de la Norma, concerné par ce projet. L'implantation d'une nouvelle ZSC entraînerait un grave déséquilibre trop exiger du territoire Mauriennais conduira à défaire tout ce qui a été mis en oeuvre ces dernières années, tant par les élus locaux que par l'État pour le rendre attractif et dynamique. Aussi, Monsieur le Ministre, je souhaite connaître les intentions réelles du gouvernement sur ce projet et sur son dimensionnement avoir des éclaircissements sur les impacts prévisibles et savoir quelles alternatives à l'exploitation de nouvelle carrière de ce type ont été étudiées dans d'autres régions du territoire national. Je vous remercie. Merci monsieur le ministre. Monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Berthet vous alerter sur un enjeu économique absolument fondamental. Vous avez raison, la Savoie possède un fleuron industriel avec l'usine de Placoplatre à Chambéry et cette unité de production qui rayonne sur le quart Sud-Est de la France et au-delà, est une filière d'excellence, notamment pour la transition énergétique, notamment d'ailleurs pour la rénovation des bâtiments. Cette unité d'ailleurs indispensable au maintien de l'activité nouvelle de recyclage de déchets de plâtre dont la collecte va être améliorée avec la montée en puissance d'une filière de responsabilité élargie du producteur pour la gestion des produits et des matériaux de construction. Il faut donc sécuriser l'approvisionnement en gypse pour ce site industriel unique c'est crucial, vous l'avez indiqué la vallée de la Maurienne. D'importants gisements qui sont propices à cet approvisionnement ainsi que des infrastructures qui favorise l'usage de mode durable alternatifs à la route et les atouts de ce territoire sont évidemment sans équivalent en France comme cela a été reconnu dans le schéma régional des carrières. le gouvernement a décidé en 2021 de lancer une démarche en vue d'instaurer une zone spéciale de carrière qui vise à garantir la pérennité de cette activité dans le respect de règles environnementales essentielles associer le public est apparu indispensable dans un esprit de transparence, de lisibilité, c'est la motivation de la concertation préalable qui sera lancé très prochainement par le préfet de Savoie, sous l'égide des garants désigné par la commission nationale du débat public et à laquelle je vous invite évidemment à participer participer à faire participer les résultats de cette concertation, pour répondre précisément aux demandes de calendrier que vous évoquez permettront d'affiner le périmètre exact pour cette zone spéciale de carrière au au sein de laquelle un projet pourra ensuite être autorisées après avis de l'Autorité environnementale, ce sont nos procédures l'autorité environnementale étant chargée de veiller à la conciliation des intérêts économiques fondamentaux que vous avez rappelé et de la préservation de l'environnement et de la biodiversité. C'est à l'issue de ce temps de concertation que le périmètre précis pour être prochainement défini. Je vous remercie. Si elle Madame Berthet. 12 secondes. Oui, Monsieur le Ministre, je le redis, il faudra vraiment être à l'écoute les élus Mauriennais soutenu par le conseil départemental de la Savoie sont fermement à ce opposés à ce projet trop largement dit Miss de dimensionner pardon et par ailleurs une pétition a déjà recueilli près de 10.000 signatures. Merci cher collègue. La parole est maintenant monsieur Jean Marie maison. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre à Petr en Moselle, le dispositif argent de poche, pourtant plébiscité. N'est plus d'actualité. Concrètement, afin d'être en conformité avec la règle. L'élu de ce territoire semi-rural ne peut plus proposer à des jeunes de sa commune de participer dans l'intérêt de la collectivité a des chantiers de quelques jours contre gratification les chantier et stage à à caractère éducatif ont et là c'était recentré sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il bénéficie à ce titre d'un régime d'exonération des cotisations sociales à verser à l'Urssaf. Dès lors qu'ils sentent notamment porté par des EPCI, ce qui n'est bien évidemment pas le cas d'une commune rurale dans ces conditions, les jeunes mosellans ne bénéficient pas tous des mêmes droits et force est de constater avec le maire de Petr qu'il y a manifestement ici. Rupture d'égalité et nombre d'élus locaux de demander avec lui que ce dispositif qui favorise l'engagement des jeunes et leur participation à la vie communale s'étendent bien à l'ensemble des territoires d'un territoire. Quelle que soit sa spécificité zone semi-rurale ou et rural comprise et s'applique indifféremment à tous comme prévu à l'origine. Êtes-vous Monsieur le Ministre, prêt à entendre leur requête à la la requête leur requête à laquelle je m'associe pleinement tant elle me paraît légitime. Merci, monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Mison pour répondre directement ce dispositif peut en effet être clarifiée ou évoluer mais je vous remercie de me donner l'occasion de rappeler en quelques mots, comme vous l'avez fait l'opportunité que constitue ce dispositif argent de poche pour les jeunes et les efforts du gouvernement afin de l'étendre aux territoires ruraux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les chantiers stage à caractère éducatif sont des actions mises en oeuvre à l'initiative de communes ou d'associations locales à destination le jeune sans activité ou en difficulté entre 14 et 26 ans, ils sont déployés dans le cadre du programme Ville-Vie-Vacances dont le régime social spécifique des rétributions a été pérennisé par une circulaire de l'Acoss, en juillet 2015, les sommes versées en contrepartie de ces activités sont assimilables au regard des prélèvements sociaux à des gratifications versées aux stagiaires en milieu professionnel et sont par conséquent exclues de l'assiette de cotisations à l'occasion du comité interministériel des ruralités à l'Automne 2021. L'extension de ce dispositif aux territoires ruraux a justement été annoncé et conformément à une instruction de fin 2021 du ministre des Comptes publics. Le régime social spécifique des opérations réalisées dans le cadre du programme Ville-Vie-Vacances a été autre étendue au territoire situé en dehors du périmètre des QPV notamment dans les zones rurales. Dès lors que les chantiers et stage à caractère éducatif sont agréés et comme pour ce programme ses actions devront avoir une visée citoyenne éducative, culturelle, sociale ou bien environnementale en vue du traitement des demandes concrètes d'application de ce dispositif de ce contrôle et de la clarification que vous évoquez notamment cette instruction a été diffusée et rediffusée auprès de l'Urssaf des Caisse Générale de Sécurité sociale dans les départements et les régions si des clarifications sont encore nécessaires. Nous sommes évidemment prêts à les apporter pour qu'il y ait pas de sentiment de discrimination ou de non prise en compte de ces demandes. RC monsieur Bison. Écoutez, monsieur le Ministre, moi je suis très satisfait de votre réponse. Ce que je regrette c'est qu'elle ne soit pas encore parvenu. En tout cas dans le département de la Moselle mais je me ferai fort dans. D'échanger sur ce thème avec le maire qui m'a sollicité. Merci beaucoup de votre réponse. Merci monsieur Frédéric Marchand maintenant. Si Monsieur le président, Monsieur le Ministre, je voudrais attirer votre attention sur l'explosion des tarifs de fourniture d'énergie et leur impact sur l'institution intercommunale D. Watrin. Du littoral nord de la France. Cette institution intercommunale a été créé il y a plus de 40 ans pour mettre en place et gérer les grands ouvrages d'évacuation des crues D. Watrin et notamment des stations de pompage de grande capacité. Cette situation est unique en France et s'explique par le fait que le territoire est un pôle d'air avec des Terres situées en dessous du niveau de haute mer, à l'instar de ce qu'on connaît aux Pays-Bas ou en Flandre belge ces installations consomment en période de crue, essentiellement en hiver de fortes quantités d'énergie pour protéger 450.000 personnes des biens et des activités agricoles, industrielles et commerciales importantes contre les inondations sur un périmètre de plus de 1000 m2 dans un triangle regroupant Saint Omer Calais et Dunkerque. La mobilisation des pompes se fait en application du protocole de gestion approuvé par arrêté préfectoral et les dépenses effectives très variable d'une année à l'autre en fonction des conditions hydrométrie qu'ces dépenses pèsent très lourdement sur le budget de l'institution en 2022 avec l'application des nouveaux tarifs les dépenses se maintiennent à hauteur de celle de 2021, mais en ayant pompé que 30% du volume de l'année précédente. Elle se serait élevé à plus de 2 millions sur la base de la même consommation pour un budget de fonctionnement de 3 3 millions huit cette situation est très préjudiciable pour l'institution qui doit en outre réalisé d'importants investissements dans le cadre du programme d'action de prévention contre les inondations du Delta de la pour pour maintenir en état un parc d'ouvrages vieillissants et se préparer à faire face aux conséquences du changement climatique. Par ailleurs, il est à noter que la réforme de la compétence Gemapi a fortement alourdi la fiscalité sur la population locale. Au vu de ces différents éléments. Il apparaît urgent de trouver des solutions qui puissent permettre à l'institution de continuer à assurer sa mission de protection du territoire et de ses habitants contre les inondations aussi. Je vous demande d'étudier la possibilité que cette institution puisse bénéficier de mesures exceptionnelles en particulier du bouclier tarifaire afin de limiter l'impact de l'augmentation du prix de l'électricité sur son budget et ainsi pérenniser ces actions au service du territoire. Merci. Merci monsieur le ministre. Monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, marchant, vous évoquez la situation dans un contexte de coût de l'énergie que nous savons élevé de l'institution intercommunale d'Éva tringle du littéral nord et plus particulièrement les conséquences de cette hausse des tarifs sur son budget. Dans un contexte où celle-ci gère notamment des stations de pompage de grande capacité pour faire face à l'augmentation sans précédent des prix de l'électricité, l'institution communale ta soutenance d'institutions intercommunale des. Comme les autres collectivités ou leurs groupements de même taille bénéficie de plusieurs dispositifs de soutien spécifique mise en place par le gouvernement en 2023, le niveau de la part d'assises sur l'électricité, l'ex-TI CFE est maintenu au minimum communautaire pour tous les consommateurs, sauf ceux qui bénéficierait déjà de taux très réduit ou d'une exonération pour l'institution intercommunale des Vatrin la baisse du niveau de l'A6 sera de 50 centimes d'euros par MWh prolonger tout au long de l'année 2023. Le gouvernement a aussi prolongé cette année le bouclier tarifaire sur l'électricité pour les plus petites collectivités l'institution intercommunale des Éva train de là aussi dans le budget excède ce critère ne peut pas bénéficier de ce bouclier directement mais elle est en revanche éligible à l'autre dispositif, c'est que c'était un peu complexe l'amortisseur électricité qui est mis en place depuis le 1er janvier de cette année pour aider précisément les collectivités qui ne sont pas directement éligibles à un dispositif de bouclier concrètement l'état prend ainsi en charge 50% du coût de l'appart énergie hors taxe au-delà d'un prix de référence de 52, 180 euros par MWh dans la limite d'une part énergie de 500 euros par MWh, mais le seuil à retenir c'est bien c'est 180 euros et cette baisse de prix apparaîtra directement sur la facture des consommateurs ou des collectivités concernées avec une compensation financière versée par l'État aux fournisseurs d'énergie pour bénéficier de cette aide, il n'y a qu'une seule démarche à faire, c'est remplir l'attestation d'éligibilité en privilégiant évidemment les recours au système en ligne l'attestation. Que déjà l'immense majorité des fournisseurs, a mis en place si vous souhaitez que nous étudions en plus en plus de détails. Le situation particulière de l'institution intercommunautaires. Je suis à votre disposition avec mes collègues. Pour ce faire. Merci, monsieur le Ministre, la parole est à madame Muller-Bronn. Merci monsieur le président, Monsieur le ministre, ma question porte sur l'insuffisance de rotation des locataires dans le parc social et les difficultés rencontrées par les maires pour procéder à de nouvelles attributions de logements. Il s'agit de locataires entrée dans le parc social à une époque où il remplissait les critères de revenus et de situations de familles logées pour certains dans des appartements de grande surface avec un loyer très modéré. 20 ans plus tard, leurs revenus ont augmenté, où les enfants sont partis, et ils ne sont plus éligibles à du logement social. Et pourtant, ils restent dans leur logement. Cette situation contribue à aggraver la pénurie de logements pour des ménages modestes qui eux devraient pouvoir y accéder. J'ai l'exemple à Obernai dans mon département d'un élu membre d'une scène qui m'explique que sur un parc de 756 logements. Il y a 400 dossiers en attente, et seulement 40 appartements libérés par an. À ce rythme, on en a pour 20 ans et autant de pertes financières pour les collectivités puisque ses loyers ne sont pas réactualisé. Les maires ont également alerté sur un phénomène hélas répandue. Ils savent très bien que parmi ses locataires. Certains sont eux-mêmes propriétaires de logements qu'ils louent sur le marché privé. Monsieur le Ministre, il faut faire évoluer la loi. L'expulsion n'étant pas une solution, soit les personnes dont les revenus sont largement supérieur au barème accepte de libérer leur logement au bénéfice bien sûr de ménage jeune modeste soit pour des raisons d'attachement à leur lieu de vie, ils peuvent rester dans leur logement en acceptant une augmentation proche du marché privé. Face à la pénurie de logements aux factures énergétiques et aux obligations de rénovation thermique qui incombe au bailleur. Il est urgent de lutter contre les abus. Merci. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Muller-Bronn vous alerter sur les enjeux relatifs aux situations de de sous occupation et l'importance d'améliorer la mobilité résidentielle, convient de préciser que le phénomène de sous-. Occupation du parc social est très important c'est vrai, mais moins importants que dans l'ensemble du parc de logements et ainsi 46% des ménages locataires du parc social sont en situation de sous-peuplement contre 71% pour l'ensemble des Français. Le traitement de cet enjeu nécessite des actions législatives parfois de long terme, vous l'avez dit, qui s'appuie tant sur la production que sur les attributions de logements sociaux l'apporte ainsi une action forte sur la restructuration de l'offre ayant permis notamment dans le cadre du plan de relance de traiter près de 50.000 logements afin d'ajuster leur typologie aux besoins du marché local de l'habitat, c'est une des. Deux autres des orientations de la réponse. De plus, le développement de produits intermédiaires comme le bail réel solidaire ou le logement locatif intermédiaire est une voie d'amélioration importante pour cette mobilité dans les parcours résidentiel sur les attributions elle-même en cas de sous occupation du logement depuis la loi Elan, le bailleur doit proposer aux locataires. Un nouveau logement correspondant à ses besoins dans les zones géographiques qui sont caractérisés par un déséquilibre important entre offre et demande de logement, les locataires qui sont dans cette situation auront refusé et qui aurait refusé 3 offres de logements de relogement perdent leur droit au maintien dans les lieux. Cela ne s'applique toutefois pas aux locataires âgés de plus de 65 ans ainsi qu'aux locataires qui présenteraient une fragilité particulière. Cela est normal et protecteur. Il faut aussi souligner une importante évolution en cours c'est la gestion dite en flux des logements sociaux qui permet au bailleur de s'affranchir des périmètres de programmes et le contingent qui touche les logements locatifs sociaux. L'analyse des impacts de ces mesures qui sont souvent récente pour conduire le gouvernement à envisager, a proposé le Parlement a proposé aussi ou à adopter le cas échéant, des évolutions législatives de ces dispositifs piloter localement. C'est un chantier que nous sommes prêts avec le ministre chargé du logement à examiner avec. Oui madame Muller bonne 13 secondes. Monsieur le Ministre, je vous remercie. Ces problématiques représente 1 à 2% du logement social, mais sur tout le pays. C'est vrai que. Ça ça libérerait ça permettrait aux mères de mieux accueillir des des primo-accédants au logement. Merci. Merci, cher collègue, la parole est maintenant monsieur Olivier Cigolotti. Merci monsieur le président, Monsieur le ministre, ma question concerne le contrôle technique obligatoire pour les deux-roues motorisés. Le compromis telle qu'il est formulé dans la directive relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur laisse à chaque pays l'opportunité d'introduire ou non un contrôle technique périodique pour les deux-roues roues motorisés suivant le principe de subsidiarité en France un travail a été menée sur les dispositions de la directive qui permet aux États membres de déroger à son application en proposant des mesures alternatives bien plus propice à améliorer non seulement la sécurité mais également la performance environnementale de ces véhicules. Ces mesures alternatives couvre tout le spectre des enjeux auxquels sont confrontés ces véhicules permis équipements de protection, renforcement des plans départementaux d'actions de sécurité routière infrastructure routière, respect des normes de bruit limitations de vitesse prime à la conversion zones à faibles émissions ces dernières sont proposées par le gouvernement en collaboration avec la Fédération des motards. Pourtant, Monsieur le Ministre, le 31 octobre 2022. Le Conseil d'État a remis en cause cette orientation du gouvernement arguant que ces mesures étaient insuffisantes et que l'ambition environnementale était insatisfaisante. Alors que la directive ne formule strictement aucune exigence pour les deux-roues motorisés par ailleurs les études les plus récentes et détaillé monte que moins de 0 5 % des accidents de deux-roues motorisés sont liés à un problème sur le véhicule. C'est pourquoi le contrôle technique obligatoire ne semble absolument pas constituer une mesure P1 pertinente alors qu'une baisse de 19% de la mortalité à deux-roues motorisés est enregistrée depuis 10 ans et que les mesures alternatives reste bien plus adapté aux aux objectifs poursuivis. J'aimerais connaître Monsieur le Ministre, comment le gouvernement compte continuer le travail engagé sans imposer un contrôle technique obligatoire et contraignant pour les deux-roues motorisés, je vous remercie. Si Monsieur le Ministre. merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Cigolotti vous touchez du doigt problématique sensible qui. Prend un certain temps depuis mon arrivée au ministère des Transports où sans rappeler tout l'historique, vous l'avez indiqué brièvement une directive de 2014 prévoit soit l'imposition d'un contrôle technique, soit des mesures alternatives avec une optique de sécurité routière puisque, il y aura plusieurs objectifs possibles, c'est l'optique qui a été alors retenu la vérité m'oblige à dire aussi, parce que cela a été rendue publique par la Commission européenne que sans doute un nouveau projet de directive ou de règlement européen sera dans les prochains mois proposée et qui très certainement cette fois imposera un contrôle technique pour les deux-roues sans mesures alternative possible dans le cadre juridique actuel, le gouvernement a, comme vous l'avez souhaité ou souligné. Préféré développer concertée des mesures alternatives au contrôle technique dont on pensait qu'elle pouvait atteindre comme prévu par la directive d'ailleurs les mêmes objectifs. Ce travail a fait l'objet de plusieurs étapes d'un décret à l'été 2021 qui devait imposer le contrôle technique qui a été ensuite abrogé pour travailler de nouveau sur des mesures alternatives ce travail a été conduit par mes prédécesseurs notamment et vous l'avez dit, le 31 octobre dernier le Conseil d'État a indiqué que les mesures proposées n'étaient pas suffisantes et je cite les termes du Conseil d'État. Il a indiqué que de telles mesures ne peuvent être regardées comme trop comme trop 4 comme trop ponctuels et manifestement insuffisantes pour assurer efficacement la sécurité des usagers au regard des statistiques pertinentes de sécurité routière pour le dire très clairement, la décision du Conseil d'État ferme la voix des mesures alternatives aujourd'hui et imposera la mise en place d'un contrôle technique. C'est dans cette optique, bien que ce ne soit pas l'option qu'avait retenu le gouvernement initialement que j'ai engagé un travail de concertation avec les associations de motards, les autres associations également je serai amené à présenter dans quelques semaines le résultat de cette concertation. Je le dis très sincèrement, nous aurons à mettre en oeuvre un contrôle technique mais je souhaite qu'ils soient respectueux de ses équilibres et nous aurons à tirer toutes les conséquences de cette décision de justice, après avoir fait tous les efforts nécessaires pour que les mesures alternatives puissent vivre mais ces nouveaux le nouveau cadre juridique qui devra être respectée à l'issue de la décision du Conseil d'État.

c'est-à-dire en privilégiant un contrôle principalement tourné sur le le niveau des émissions sonores et polluante et peut plus particulièrement pour les cyclomoteurs de moins de 50 cm3. Merci la parole est maintenant madame Sylviane Noël. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, je souhaite attirer votre attention sur la situation que traverse les infirmiers libéraux suite à une décision de la CPAM de Haute-Savoie de modifier les les modalités de remboursement de leurs indemnités kilométriques depuis le mois de novembre dernier qui pénalise fortement les infirmiers exerçant en zone de rurales et de montagne. Car oui, dans ces secteurs parfois éloignées difficiles d'accès escarpé enneigé. Une bonne partie de l'année, le rythme de visite des patients est fortement différent de l'exercice en milieu urbain et de fonds de vallées. Ces contraintes doivent être prises en compte dans le calcul des compensations kilométrique, faute de quoi le manque à gagner pour les infirmières est inévitable. Ainsi la différence entre le nouveau calcul et et l'ancien mode de calcul est stupéfiante. À titre d'exemple, sur la commune de Passy là la perte de revenus s'élève à 23% au Grand Bornand à 15% et atteint à 22,6%. Le manque à gagner est réel et se produit dans un contexte pardon d'inflation fort qui touche particulièrement les carburants ces infirmiers libéraux réalise au quotidien un travail exceptionnel au plus près des patients et des territoires permettant le maintien à domicile et contribuant ainsi au désengorgement de nos établissements de santé fortement en Bolivie par la pénurie de personnel inédite que nous connaissons. Aussi, je souhaiterais connaître les mesures que vous avez envisagé de prendre pour remédier à cette injustice. Je vous remercie. Merci beaucoup monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Noël je partage avec vous la nécessité de prendre un peu de sirop et je répondrai néanmoins au nom également de mon collègue ministre de la Santé François Braun. Le coût des transports de manière générale est évidemment au coeur des préoccupations actuelles de nos concitoyens et c'est particulièrement vrai pour un certain nombre de professionnels dont les infirmiers libéraux qui, par définition, se rendent au domicile des personnes qu'elles aident et soigné. En 2019, les partenaires conventionnels avait justement convenu d'un abattement du tarif de remboursement des indemnités kilométriques au regard de la distance journalière facturé par l'infirmier. Cette nouvelle disposition importante permet de limiter les indus et de laisser la possibilité de facturer comme on le dit en étoile, c'est-à-dire sans mesurer à chaque fois la distance entre le domicile du patient et le cabinet de l'infirmier ou d'infirmière et dans un esprit de souplesse avait été laissé la possibilité d'adapter les modalités de facturation aux spécificités locales. ce cadre et dans cet esprit qu'un nouvel accord de la CPAM de Haute-Savoie mettait en place met en place, toujours des règles plus avantageuses avec une prise en compte des kilomètres effectués au sein d'une même commune à partir d'1,5 kilomètres kilomètres qui n'était auparavant pas indemnisés et une valorisation des indemnités au titre de la zone de montagne, étendu à tout le territoire du département de la Haute-Savoie, de manière plus globale. Le gouvernement soutient l'implication des infirmiers libéraux dans la prise en charge des patients à domicile avec un avenant du mois de janvier dernier pour le doublement des nouvelles rémunérations sur le bilan des soins infirmiers sur la période qui va jusqu'à 2024 2024 ça représente plus de 200 millions d'euros. Des mesures qui s'ajoute aux dispositions d'un avenant de 2019 améliorant la prise en charge et l'accès aux soins des patients et dans le budget de la finance de la Sécurité sociale. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023. Celle-ci confie de nouvelles missions aux infirmiers comme élargissement de leurs compétences vaccinales ou une expérimentation pour la réalisation de certificat de décès qui est de nature aussi améliorer le pouvoir d'achat, pour être très concret sur la question des indemnités en particulier et pour prendre en compte des situations locales, nous sommes prêts avec François Braun a regardé chaque situation avec vous dans les prochaines semaines. Merci madame Noël. Merci, monsieur le Ministre pour. Votre exposé, j'entends ce que vous me dites mais sur le terrain, les infirmières ont une toute autre vision de ce qui se passe. 14 euros 28 pour 24, visite, soit 60 centimes en moyenne d'indemnités horokilométrique montagne par visite. Voilà la réalité de ce que vivent les infirmières dans certains secteurs de Haute-Savoie. Croyez-moi à ce niveau-là de revenus, on ne peut pas survivre. Et je pense que c'est un le genre d'économies de bouts de chandelle qui malheureusement ne nous mènera à rien ne nous mènera qu'à de voir. Entraîner des patients à être réhospitalisé ou ne plus être maintenues à domicile, et ça nous coûtera beaucoup plus cher au final qu'il y a un réel risque de pénurie d'offre de soins dans ces secteurs vraiment il y a urgence. Merci. Merci cher collègue. La parole est maintenant Madame Victoire Jasmin. Merci monsieur le président, Monsieur le ministre, ma question porte sur le Conseil pour les droits et devoirs des familles en outre-mer c'est un dispositif d'aide à la parentalité fondée sur l'action sociale et éducative facultatif faut toutes les communes depuis la loi dite engagement et proximité.

c'est peut être également un outil pour les mères. Chaque fois que le comportement d'enfant entraîne des troubles à l'ordre et à la sécurité publique. Or, dans ce contexte croissant d'insécurité. Les élus locaux d'outre-mer sont inquiets en effet les chiffre fourni en 2021 par le ministère de l'Intérieur font figure et les départements d'outre-mer parmi les plus criminogènes en France, la population en Guadeloupe mais aussi en Guyane et à Mayotte se retrouvent souvent. Beaucoup plus d'ailleurs qu'Hexagone confronté à des actes de vols et de violences volontaires. Sur l'année 2020. La Guadeloupe. En Guadeloupe, les infractions des mineurs en matière de sécurité. Pose problème. Les problèmes également la sécurité routière. Les problèmes de stupéfiants les infractions en lien à la conduite sans permis. Si Tristan Si Tristan cette insécurité concerne également les mineurs d'après l'enquête virage de 2018 dans les outre-mer il en ressort également une fréquence plus élevée des violences intrafamiliales que dans l'Hexagone. Par ailleurs, la Guadeloupe est confronté à un phénomène de bandes organisées. Et à un niveau de délinquance juvénile important dès lors la prévention de la délinquance par des actions de sensibilisation complétant s'est déployée en milieu scolaire est fondamental pour impliquer aider les familles en difficulté. Il convient de permettre aux élus locaux d'activer tous les leviers en matière de sécurité, notamment au sein des groupements locaux de prévention des ici et le SPD des SPD mais aussi par la généralisation des conseils pour les droits et devoirs des familles. Je souhaite Monsieur le Ministre, que vous puissiez nous permettre de généraliser ce dispositif. Est-ce que c'est possible selon vous. Merci. Merci pour voir et prendre la parole est à monsieur Jean-François Carenco, ministre délégué chargé des Outre-mer. Le président. Madame la sénatrice. Comme vous le savez, les maires et vous l'avez dit, ont des fonctions essentielles, en matière de prévention de la délinquance sur leur territoire. Ils jouent en effet un rôle prépondérant dans le diagnostic des phénomènes de délinquance dans les actions de prévention à mettre en oeuvre. On a un public parfaitement identifiés. Par ailleurs, une partie pleinement la dynamique locale que les préfets doivent impulser. Des des préfets de département doivent impulser dans le cadre du plan départemental de prévention de la délinquance qui décline la stratégie nationale en la matière. Dans l'exercice de ses missions, le maire dispose de nombreux outils réglementaires dont le rappel à lors de la transaction le con et le Conseil des droits et devoirs des familles c'est d'EDF qui fait l'objet de votre question. L'ensemble de ces dispositifs doit permettre aux maires d'agir efficacement à l'égard des mineurs en situation de fragilité comme et l'égard de ceux qui sont déjà passés à l'acte et qui courent le risque d'un basculement définitif dans la délinquance. Lieu de coordination des dispositifs de prévention. Le CDF. Est également un espace de dialogue et d'alerte pour tous les jeunes concernés, une intervention de l'autorité républicaine incarnée par le maire, en présence des parents et il me semble-t-il de nature à faire prendre conscience à chacun de ses droits et devoirs. Le CDD F. Offre effectivement un cadre juridique sécurisé où le maire peut recevoir le jeune mineur sa famille revenir sur le fait produit dans la commune a rappelé ses parents toute la à ses parents toute l'importance de leur rôle éducatif. De la sorte le CDF permet d'assurer la prise en compte et le traitement des faits commis sans avoir. À solliciter une réponse judiciaire dé facto limitée par la minorité de leurs auteurs. Les parents sortent. Responsabilisés confortés dans leur rôle. Prise en compte. Le jeune. Se sont considérés individuellement dans son parcours et le maire joue alors pleinement son rôle de proximité auprès de la population par le, par laquelle pour laquelle il a été élu. Je comprends donc parfaitement votre opinion sur l'importance d'essayer Il faut encourager les maires de chaque commune à mettre en place et tout outil réglementaire. Laissés à leur disposition. Suite à votre question, je saisirai directement les préfets pour qu'ils impulsent auprès des maires. La nécessité de réunir ses instances. Par ailleurs, le ministère de l'Intérieur des Outre-mer a sollicité le secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation pour qu'il se rapproche de l'Association des maires de France étudie avec elle comment promouvoir efficacement ce dispositif nous allons le faire aussi à notre niveau au cas par cas. Je précise aussi l'expérience du préfet Lalanne qui est en Martinique. Et ministre vous avez largement dépassé votre temps. Merci, merci de respecter le temps pour les questions suivantes. La parole est à monsieur Yves Détraigne. Merci monsieur le président. Monsieur le Ministre, j'appelle votre attention sur ma question du premier avril 2021. Contrairement à ce que la date pourrait le laisser croire, ce sujet très sérieux qui porte sur la pension alimentaire et concerne des millions de familles auraient mérité une réponse du gouvernement la création d'un barème a permis de simplifier le calcul de la pension et il est normal qu'il figure sur le site de la chancellerie. Mais attention à ne pas vouloir trop simplifier les choses, car les enjeux sont importants. D'abord, il serait bon de préciser si sur le site que le barème n'a qu'une valeur indicative. Ceci est d'autant plus importante que ce barème. Propose un montant de pension à verser en cas de résidence alternée. Or, dans 75% des divorces qui fixe une résidence en alternance aucune contribution alimentaire n'est prévue. Même indicatif. Se paraît bleu officiel sans notice explicative peut induire en erreur. Plus étonnant encore la le barème laisse laisse que les ressources du parent bénéficiaire du versement ne sont pas prises en compte dans le calcul de la pension. Ce qui est contraire aux dispositions du code civil. Monsieur le Ministre, il ne faut pas sacrifier la justice familiale sur l'autel de la simplification voire de la des jus dire. Six rations vous avez bien compris du contentieux familial, pouvez-vous nous va apporter clusse et éclaircissements utiles. Merci, monsieur le Ministre. Monsieur le président, monsieur le sénateur, de train. Le gouvernement est pleinement mobilisé dans cette lutte active contre retard et les impayés de pensions alimentaires. J'ai réussi, j'ai reçu hier pour une réunion de travail. Le directeur général de la CNAF qui doit travailler qui va prendre en charge à terme les c'est la CAF qui vont prendra à terme en charge le versement des pensions alimentaires. J'en veux aussi pour preuve. La récente systématisation de l'intermédiation financière des pensions alimentaires par la CAF donc qui réduit fortement les inquiétudes liées à la prise en charge financière de l'enfant. Nous progressons sur le sujet et je réunirai bientôt tous les directeurs de CAF en accord avec le directeur général de la CNAF et en 1er lieu, je vais vous rassurer le caractère purement indicatif purement indicatif. Vous l'avez dit figure au moins à deux endroits sur le site internet d'une part dans la fiche intitulé tout savoir sur la pension alimentaire. D'autre part, dans le mode d'emploi du simulateur. En 2ème lieu bien évidemment la résidence alternée n'exclut pas par principe le versement d'une pension alimentaire en pratique une telle versée dans 2 hypothèses, lorsque les parents ne s'entendent pas pour partager les frais d'éducation et d'entretien de l'enfant. mieux quand lorsque l'un des parents ne peut assumer la charge financière de la résidence alternée. La résidence alternée ne peut donc pas être exclus du barème qui je le rappelle est strictement indicatif. En 3ème lieu, je rappelle que la pension alimentaire est déterminée par le juge qui prend en compte les revenus et les charges de chacun des parents. Il n'y a qu'un objectif, assurer l'éducation et l'entretien de l'enfant. En outre, je précise que la circulaire du ministre de la Justice du 12 avril 2010 qui accompagnaient la diffusion juridiction de la de référence. Cette table et déterminé sur la méthode dite du pourcentage des revenus qui consiste à appliquer au revenu du parent débiteur hein Kofi en correspondant au coût relatif de l'enfant. Cette méthode produit des résultats identiques à la méthode dite du partage pour les revenus inférieurs à 5000 euros, c'est-à-dire dans le sens de l'application de la table. Cette méthode cinq produit des résultats identiques à la méthode dite du partage des revenus fondée explicitement sur le revenu des deux parents ainsi les informations diffusées sur le site internet qui sont seulement destinées à permettre le bon fonctionnement de la table et du simulateur ne me semble pas ils ne me connaissent pas les règles du code civil sur la détermination des pensions alimentaires. Mais le sujet est à l'ordre du jour dans toutes les cas. C'est. Monsieur Détraigne 12 secondes. Merci Madame, Sonia de la Provoté. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre. Je souhaite attirer votre attention sur l'incertitude qui entoure le régime juridique des colocations de seniors. Le code de l'action sociale et des familles prévoit que les les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les études sont des établissements qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apporte à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale. Ce même code prévoit la création que la création de cet établissement est soumise à une autorisation délivrée, soit par le président du conseil départemental, soit par le directeur de l'ARS ou conjointement. La colocation seniors se développent comme alternative à l'entrée, on n'est pas des permet de rompre l'isolement social. C'est une demande forte du public visé et des familles. En effet, la colocation apporte aux usagers un cadre vit sécurisant avec des prestations, telles que la présence permanente de personnel des espaces de vie communs mutualisés cuisine salon et Cependant, elle propose ou impose des prestations hôtelières. Forfait forfaitairement aux résistants sans aucun cadre prévu, restauration, ménage, gardiennage. Et gestion de des ressources humaines et des auxiliaires de vie. Ces structures ressemblent fort à des établissements médico-sociaux et de Redon devrait donc être soumis à une autorisation ou du moins un cadre or face à un flou juridique certains certains ont ainsi ouvert leurs portes sans avoir eu près au préalable obtenu l'autorisation de création auprès des autorités compétentes. dans ces circonstances, dit le président du conseil départemental, ni le directeur général de l'ARS ne peuvent procéder aux vérifications nécessaires et de base pour s'assurer, avant l'ouverture que les conditions d'accueil des personnes âgées notamment les qui les questions de conformité sont garantis. Ainsi, Monsieur le Ministre, de quel régime juridique relève ses structures et quelles sont leurs obligations pour obtenir une autorisation de création des évolutions réglementaires sont-elles envisagées pour clarifier le statut de ces structures et permettre un meilleur contrôle de certains débordements. Je vous remercie. Monsieur le président, madame la sénatrice la définition générale de la colocation remonte. Ah, la loi du 6 juillet 1989 qui a décrit comme la location d'un logement par plusieurs locataires constituant la résidence principale et faisant l'objet d'un ou plusieurs contrats entre les locataires et les bailleurs. Il s'agit là des dispositions de droit commun. Qui ne relèvent pas du code de l'action sociale et des familles les habitats que vous évoquez. S'adressant aux personnes âgées en perte d'autonomie et proposant différents services s'apparente en effet davantage à des résidences services seniors. comme telle, elle ne font pas l'objet d'autorisations médico-social car elle ne propose, outre le logement que les prestations hôtelières et d'aide administrative. Vous faites le constat. Que les autorités compétentes sur le Champ de l'autonomie que sont le président du conseil départemental, le directeur général de l'ARS ne sont pas en mesure, c'est vrai de procéder aux vérifications nécessaires dans la préalables dans la mesure où ces colocation ne sont pas des établissements médico-sociaux. Cependant, bien que la réglementation, je le confirme ne pas de contrôler en colocation des inspections sont cependant envisageable dans les cas suivants, tout d'abord lorsque les services départementaux comme l'ARS. Ont toute autorité pour assurer un contrôle auprès d'un service d'aide et d'accompagnement de soins infirmiers à domicile qui eux font l'objet d'autorisation intervenant auprès des colocataires. Le préfet peut lui aussi intervenir. Immobiliser les agents de contrôle de l'ARS, ainsi que des autres services de l'État au motif de contrôler les services sociaux médico-sociaux sociaux intervenant par ailleurs. Auprès des colocataires, quelle que soit l'autorité de tutelle. Enfin, les services des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités peuvent intervenir dans le Champ de la protection des consommateurs par rapport aux prestations Frac facturés. Au 4h par les services sociaux ou médico-sociaux précités intervenant à leur domicile. Vous le voyez le développement d'alternatives à l'Epad, puisque c'est ça. Ce dont il s'agit, ne fait pas l'objet d'autorisations préalables. Mais de ce fait pas non plus en dehors de tout contrôle et ministère des solidarités pleinement mobilisés pour garantir la plus grande qualité de l'accueil d'tu es pas niemand. À toutes les personnes âgées de notre pays et effectivement ce système se développe. Et les contrôles doivent se multiplier mais ils seront à posteriori parce qu'ainsi la loi et le règlement. Merci. La parole est à madame. Monique Lubin. Merci monsieur le président, Monsieur le ministre, ma question s'adressait au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et concerne l'enjeu du développement des résidences de répit partagé lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2023, le Sénat a adopté à l'unanimité l'amendement que je portais au nom de mon groupe, afin de permettre à l'accompagnement dès 2023 du développement de 10 résidences de répit partagé sur tout le territoire français. Cet amendement a été balayée par le gouvernement ce qu'il a recouru à l'article 49.3. Nous le déplorons car ces résidents se sont, terme mixte associant des prestations hôtelières et de tourisme de qualité à la présence de professionnels médico-sociaux, nous en avons besoin sur tout le territoire, il y a en effet plus de 11 millions d'aidants familiaux en France et cette dans sur 10 refusent l'idée d'un placement définitif de leurs proches, aidés ils aspirent à ce qu'un droit au répit. Soit effectif, plus d'une dizaine de territoires et au 1er chef leurs conseils départementaux en lien avec les associations représentatives des personnes et des aidants sont ainsi porteur de tels projets et singulièrement dans les Landes co-par l'État et les départements. Ces résidences nécessite un engagement sociétal fort et spécifique de la part de l'État au titre des crédits médico-sociaux au regard du faible coût pour lui de cette mesure en regard de ce qu'elle est susceptible d'apporter à la population et aux territoires. Il nous semble légitime qui s'investissent résolument dans cette démarche et si Monsieur le Ministre des Solidarités de l'autonomie des personnes handicapées m'a signalé au cours d'une audition en commission des affaires sociales qu'il y a dans ce Plfss des crédits qui peuvent bénéficier aux porteurs de projets de cette nature. Cela n'est cependant pas à hauteur de l'enjeu aucun crédit ne semble fléchés pour ces dispositifs pour les agences régionales de santé. Je vous demande donc, Monsieur le Ministre, si le gouvernement compte mettre ces crédits à disposition. Merci, monsieur le Ministre. La sénatrice la stratégie agir, agir pour les en 2022 1022 a permis de poser le soutien aux aidants comme une priorité. Cette première stratégie comprenait parmi les 6 priorité l'ambition d'accroître et diversifier les solutions de répit. Elle était soutenue par un budget cumulé sur l'ensemble de la stratégie de 105 millions d'euros. Le gouvernement a bien évidemment la volonté de poursuivre le soutien aux aidants et a annoncé début octobre 2022 qu'une deuxième stratégie dans sera élaboré au cours de l'année 2023. Une concertation des acteurs pour la construction de cette stratégie est en ce moment conduite par le même gouvernement sous l'autorité du ministre compétent. Pour construire cette stratégie. Le gouvernement s'appuie notamment sur le rapport publié la semaine dernière par l'IGAS sur le cadre juridique et le financement du répit en parallèle la Haute Autorité de santé a été saisie sur la définition du répit et l'élaboration des bonnes pratiques professionnelles professionnels sur les actions de répit. Les auteurs recommandent de diversifier les solutions de répit notamment n'adaptant l'offre d'accueil temporaire et en améliorant l'accès au relais. À domicile et à l'accès au séjour vacances. Leurs recommandations ne vont pas dans le sens d'un déploiement généralisé des maisons de répit ou des résidences de répit partager ses modèles existants. Doivent être complétées en effet par une offre plus diversifiée de proximité accessibles, notamment le soir et le week-end. Il s'agit tout à la fois de renforcer les plateformes de répit existantes et de développer une meilleure suppléance au domicile des personnes des c'est le modèle. Vous avez cité et qui se déploie par exemple à Mont-de-Marsan avec une maison d'accueil temporaire pour les personnes âgées qui permet de l'hébergement temporaire dans une limite de 90 jours mais aussi les prises en charge ponctuelle sur la journée. Il y a l'accueil de jour, c'est en travaillant sur ces solutions adaptées diversifiées au besoin de chacun que nous pourrons assurer un meilleur soutien aux aidants qui occupe une place essentielle effective dans notre politique de solidarité. Toutes les études sont en cours en 2023 et j'espère que nous réussirons. Merci madame Lubin. Alors je, j'espère que j'ai mal compris mais si j'écoute bien votre réponse, je crois que vous m'avez dit non. Voilà donc j'espère que ce n'est pas ça. Mais non mais je, je vous ai entendu dire que vous avez parlé des maisons de répit. Vous aviez dit qu'il y en avait assez et que c'était pas la solution. J'espère que j'ai mal compris, Monsieur le Ministre. Ah non, on n'avait pas le droit. Monsieur le Ministre, non non et ici c'est pas le bazar c'est le Sénat. La parole est maintenant à monsieur Christian Klinger. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre. Depuis plus d'un. Depuis près d'un siècle, l'Alsace et la Moselle sont en partie régis par un droit local qui constitue un modèle de différenciation territoriale du droit. Produit de l'histoire mouvementée des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Le droit local alsacien mosellan et depuis 2011 un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Cela étant, au-delà de cet aspect constitutionnel le droit local alsacien mosellan règlement de nombreux aspects de la vie quotidienne et nos concitoyens, ils sont fortement attachés. Pourtant, il semblerait que l'administration centrale oublie ses particularités dans ses instructions et circulaires, notamment en ce qui concerne les jours fériés et chômés. La durée annuelle du temps de travail des fonctionnaires territoriaux a été fixé à 1607 heures. À ce sujet le code général de la fonction publique on ne peut plus clair. Il prévoit pour les agents de la fonction publique territoriale de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin que le vendredi Saint et la Saint-Étienne sont férié et chômé. Pour le calcul de la durée du temps de travail de ses agents de la fonction publique territoriale. Il y a lieu de tenir compte de ces deux jours fériés et chômés c'est-à-dire prévoir un temps de travail annuel 2593 heures et non 1607, autrement dit il n'est pas concevable que ces agents soient tenus de rattraper les heures de travail pour ces deux jours. Ainsi, Monsieur le Ministre, je me demande de bien vouloir préciser votre position sur ce sujet. Votre position est attendu par l'ensemble des agents des collectivités territoriales d'Alsace et de Moselle et par les élus locaux et ainsi vous pourrez nous rappeler votre attachement au droit local alsacien mosellan. Merci de faire la question et la réponse. Chers collègue, la parole est à monsieur le ministre. monsieur le ministre. Évidemment c'est le sénateur afin d'harmoniser la durée. Du temps de travail au sein de la fonction publique territoriale mais également avec la fonction publique de l'état de la loi de transformation de la fonction publique à supprimer. Les régimes de travaux vas dérogatoire mises en place avant 2001 dans les collectivités territoriales. Dans les délais prévus par le législateur. Les collectivités territoriales concernées sont tenus de définir dans les limites d'un an à compter du renouvellement général Georges assemblée délibérante de nouvelles règles relatives au temps de travail de leurs agents. Les dispositions de la loi de transformation de la fonction publique sont applicables aux collectivités de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui soit par conséquent appliquer la durée légale annuelle du travail effectif 2000 chance 1607 heures. L'article L 31 34 13 du code du travail prévoit comme vous l'avez rappelé, que dans ces départements le vendredi Saint. Et le 26 décembre sont des jours chômés. Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle, monsieur le sénateur à l'application des 1607 heures dans ces collectivités, la durée légale du travail s'applique en effet uniformément et indépendamment du nombre de jours chômés, qu'il s'agisse du jour férié de droit commun ou des jours chômés. Propre au départements d'Alsace et de Moselle. Mon expérience outre-mer fait que je peux vous dire que le sujet est exactement le même avec des, des jours chômés et fériés très compliqué. Les collectivités territoriales et de leurs établissements publics de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ne saurait dès lors. Se prévaloir du deux jours chômés pour définir une durée annuelle du travail inférieure à 1607 heures sans méconnaître les dispositions applicables dans la matière. Par ailleurs, ces jours fériés et chômés reste non travailler dans ces départements. Je vous remercie. Hé oui Monsieur Clean guerre comme quoi 19 secondes pour dire votre mécontentement. Je dis mais oui bah oui je partage pas votre analyse, Monsieur le Ministre, vous êtes le ministre des autres maires qui ont des spécificités vous les respecter, il faut respecter le droit alsacien mosellan le vendredi Saint, la Saint Etienne sont des jours fériés ils n'ont donc pas être travailler, il faut donc il faut modifier votre décret en rajoutant de jours fériés pour les agents des collectivités territoriales d'Alsace et de Moselle. Merci d'en tenir compte. Merci Monsieur Clean guère la parole est maintenant à Madame Marie-Claude Ryan. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre il y a 8 mois dans la nuit du 20 au 21 juin, une tempête de grêle exceptionnelles et dévastatrice a touché 46 communes en Dordogne dans le secteur du Ribeira quoi. Monsieur le ministre de l'Agriculture a dépêché sur les lieux 2 inspecteurs que j'ai avec mon collègue sénateur accompagner afin de constater les dégâts d'une ampleur démesurée et frappant durement les agriculteurs, les entreprises, les collectivités et des habitants. Mardi 24 janvier dans une large unité syndicale les agriculteurs au nombre de 300 sont venus devant la préfecture de la Dordogne exprimer leur désespoir et demandé que soit débloqué des aides du fonds d'urgence, à ce jour très insuffisant et la reconnaissance du régime de calamités agricoles. La chambre d'agriculture a évalué les pertes de culture à 25 millions d'euros quand le total des aides publiques ne couvrent que 13% du montant estimé des dégâts. À ce jour 189 exploitants agricoles ont bénéficié de 1,74 millions d'euros d'aide soit 9200 euros par exploitant en moyenne ce qui est très insuffisant. Lorsque l'on sait qu'aux pertes subies, s'ajoutent les frais de remise en culture l'achat de fourrage d'aliments pour leurs élevages et la remise en état des bâtiments et du matériel agricole depuis 8 mois. C'est un territoire meurtri qui se sent abandonné les aides consenties par l'État été étant très en dessous des dégâts constatés. Il faut Madame la Ministre avoir entendu le témoignage de ces femmes et de ces hommes qui ont tout perdu et vu ses paysages dévastés pour mesurer la détresse de cette population dont toutes les maisons toujours bâchées à ce jour, garde les stigmates de cet épisode climatique, particulièrement violents cette situation exceptionnelle Madame la Ministre nécessite des moyens exceptionnels. Et c'est la raison pour laquelle je m'a prêté ce matin a invité Monsieur le Ministre de l'Agriculture à venir en Dordogne afin qu'il puisse constater lui-même l'ampleur de cette catastrophe des indemnités des indemnisations qui sont consentis à ce jour, merci. Merci pour vous répondre. La parole est à madame Olivia Grégoire Ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, vous avez la parole madame la Ministre. Merci monsieur le président, madame la sénatrice, var, alias le ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire et. Hé bien conscient de la détresse que vous mentionnez, nos agriculteurs du terroir Ribeira quoi et je commence par vous dire que je lui transmettrai dès la sortie de cet hémicycle l'invitation que vous venez de réitérer. C'est la moindre des choses. Je tiens à apporter quelques éléments de réponse dont je ne doute pas qu'il ne vous satisferont pas totalement mais sachez, je le répète, que je m'entretiendrai avec monsieur Fesneau pour. Reparler du d'un déplacement et. D'échanges avec vous ces intempéries dramatiques que vous mentionnez ne sont effectivement pas éligible au dispositif des calamités agricoles. ce sont donc des mesures de soutien qui ont été annoncés comme le dégrèvement de la. NB, mais aussi le report de cotisations sociales et la prolongation des PGE le ministre-Fesneau a également décidé, vous le savez, d'une mission du Conseil général de l'alimentation agriculture et des espaces ruraux pour qu'on évalue très précisément les dégâts et qu'on réponde au cas par cas aux agriculteurs touchés par ces phénomènes extrêmement intense. Cette mission a recommandé. La mise en place d'un fonds d'urgence de 40 millions d'euros au moins recommandations immédiatement suivi et mises en oeuvre par le ministre-Fesneau se font état, la main des préfets pour apporter une réponse rapide aux situations de très grande fragilité que vous avez mentionnées, madame la sénatrice. elles sont accordées, dans la limite d'un plafond de 5000 euros par exploitation plafond porté au montant estimé nécessaire pour aider les exploitations les plus en difficulté dans la limite du plafond des mini-miss, vous évoquez à juste titre une aide de 9200 euros par exploitant en moyenne et cela montre que nous n'atteignons pas dans bien des situations. Le plafond des minimise qui s'élève à 20.000 euros. Les situations personnelles des agriculteurs du territoire que vous mentionnez doivent donc continuer à faire l'objet d'un examen approfondi au niveau local pour trouver des solutions qui répondent à leurs difficultés. C'est donc. Le sens de la position de monsieur Marc Fesneau et j'espère que nous aurons d'autres éléments en réponse dans les prochains jours et semaines. Merci la parole est à monsieur Jean-Pierre Moga. Merci monsieur le président. Madame la ministre. Je souhaite attirer votre attention sur la situation très difficile que traversent les transporteurs routiers, du fait de l'envolée du prix du pétrole ces derniers mois, et des conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Le coût du gazole a augmenté de 36% seulement un an, ce qui représente une hausse considérable absorber. De surcroît, l'augmentation cumulée des tarifs de péage sur les années 2022 et 2023 en prenant en compte les dernières augmentations.

Je sais Madame la Ministre que vous pourriez me répondre que les prix du pétrole ont baissé ces derniers mois, ce qui est vrai. Mais ils se sont stabilisés à des niveaux bien supérieurs à ceux que nous connaissions à l'aube du conflit avec. En Ukraine. Si l'on observe ce qui se fait autour de de chez nos voisins, on remarque que d'autres pays européens ont décidé de maintenir des dispositifs d'aide pour leur secteur de transport routier dans cet esprit. Pouvez-vous nous dire quelles sont les mesures spécifiques que le gouvernement. À neuf afin de soutenir les entreprises de transport françaises face à cette hausse des prix des carburants et aux perspectives économiques défavorables pour le 1er semestre de l'année 2023. Des aides ponctuelles et exceptionnelles pourraient être mises en place et si oui, quelles en seraient les modalités les montants budgétaires ainsi que les critères de ciblage pour les entreprises éligibles à ces dernières. Je vous remercie. Merci la parole est à madame le Ministre. Merci monsieur le président, Monsieur le Sénateur, Maugars. Votre interrogation légitime sur les dispositifs de soutien aux entreprises du transport routier face hausses de prix des carburants Quitte à vous surprendre, je ne répondrai pas que. Les carburants ont à nouveau baissé, ils sont suffisamment volatiles pour qu'on ne se réjouissent pas qu'il baisse après avoir tant augmenté. En revanche, j'ai à coeur de vous rappeler. Que le gouvernement n'a, n'a. Pas attendu et a mis en place des aides il y a plusieurs mois pour permettre à ce secteur extrêmement stratégique pour notre économie de faire face. D'abord une aide forfaitaire aux véhicules. Le gouvernement a mis en place une aide forfaitaire qui s'adressent spécifiquement à nos entreprises de transport public routier qu'il s'agisse d'ailleurs de marchandises de voyageurs de sanitaires mais aussi aux entreprises de négoce d'animaux vivants. Le téléservice qui avait été mise en place permettait de s'inscrire entre le 8 avril et le 31 mai 2022. De nombreuses demandes en recours ont été déposés jusqu'au 31 août 2022 inclus. Et je tiens à vous dire, Monsieur le Sénateur Moga que les premiers paiements issus de leurs examens. Vont intervenir. Avant la fin du 1er trimestre 2023, le montant de l'aide dépend du nombre de véhicules de l'entreprise mais aussi du tonnage de ces dernières versée en une fois cette aide forfaitaire peut atteindre 1300 euros par par véhicule, auxquels s'ajoutent, pour les entreprises de transport de marchandises ou de transport public de voyageurs d'amende par ailleurs le remboursement partiel de la TICPE si elle remplit certaines conditions, conditions qui sont toutes résumé sur le site entreprendre Point service Tiret public Point FR le remboursement est calculé à partir de la consommation réelle de gasoil d'essence ou de biocarburants. Au cours d'un trimestre et le calcul du monde ont remboursé se fait sur un taux forfaitaire ou régional les montant de la TICPE pour 2023 sont dans l'attente des communiqués par la Direction des douanes et les montants des années précédentes sont toujours en vigueur combiné ces aides devraient permettre aux professionnels du transport routier, de faire face à cette crise du carburant. Je vous remercie. Merci monsieur Moga 7 secondes. La parole est maintenant à monsieur Patrice Joly. la filière de la boulangerie, ses traditions, ses savoir-faire. Il semblerait que celle-ci soit désormais malheureusement en voie d'extinction dans nos villes et nos villages affaibli depuis plusieurs mois par la concurrence des grandes surfaces qui vendent des baguettes à prix cassés mais aussi par la hausse des prix du beurre et de la farine nos artisans sont aujourd'hui frappés de plein fouet par l'explosion de leur facture de gaz et d'électricité par feu multiplie par 10 depuis l'Automne plusieurs boulangers ont déjà été contraints de fermer boutique. Acteur indispensable de la vie délité des territoires ruraux. Les artisans sont perdues et ne demandent qu'à travailler, mais certainement pas à perte. Certes le gouvernement a mis en place pour les TPE de moins de 10 salariés avec un chiffre d'affaires annuel de moins de 2 millions d'euros et ayant conclu un abonnement d'une puissance inférieure à 36 qui avait. Un bouclier tarifaire permettant de plafonner la hausse de l'électricité de 15% à partir de février 2023 jusqu'en décembre de cette année. De même, il en est de même s'agissant du gaz. Or, de nombreuses boulangeries consomme bien plus et sont donc de fait exclus du dispositif, c'est le cas notamment qu'on vient de me rapporter sur la commune de Mylène où le maire m'a indiqué effectivement les difficultés du boulanger de sa commune dans la Nièvre. Les fournisseurs ont par ailleurs accepté que l'ensemble des pays ayant signé des contrats d'électricité au cours du second semestre 2022 ne paie pas plus de 280 euros le mégawattheure. En moyenne sur les 2023 c'est bien mais ce dispositif laisse encore une fois de plus sur le bord de la route un certain nombre de commerces. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir m'indiquer si de nouvelles mesures en cohérence avec la réalité des territoires seront mises en place rapidement pour sauver ces commerces de proximité qui font vivre tous nos territoires et en particulier nos villages en participant à leur attractivité. Je vous remercie. De façon très directe a suggéré que si vous avez en main le cas d'une boulangerie. Avec des factures je suis à votre disposition. À la fin de la séance. Pour observer le cas. 33.000 boulangerie en France. Et non la baguette ne disparaîtra pas. On a suffisamment de raisons de s'inquiéter pour patients créé en plus il y a des difficultés, je ne les nie pas, mais notamment pour un tiers de nos boulangers qui sont dans le cas d'un renouvellement de contrat et qui ont été confrontés. Soyons clairs, vous l'avez dit, monsieur le sénateur, à des tarifs absolument aberrant au second semestre 2022. C'est bien pour ça. Que nous avons réagi et je ne reviendrai pas sur ce qu'on appelle le TRV des TPE, vous l'avez bien décrit le tarif réglementé de vente qui s'adresse à nos TPE et vous avez aussi bien décrit le fait que non. Nos boulangers, il n'y était pas beaucoup éligible parce qu'en réalité, ils ne sont pas vraiment à, au, au plafond de 36 kilovoltampères mais bien plus entre 70 80 90. Kilovoltampères donc je suis bien conscient du sujet Bruno Lemaire aussi la Première ministre aussi et c'est pourquoi nous n'avons pas attendu et nous avons dès la fin d'année dernière. mobiliser l'ensemble des fournisseurs pour qu'ils s'alignent sur ce qu'on appelle le tarif indicatif de la creux évalué aux alentours de 280 euros le mégawattheure. Qui sera le prix. Auquel paieront au maximum nos TPE et notamment celles qui ont signé, à des tarifs exorbitants. Nous avons donc ramener. Les les tarifs aberrants à un tarif quasiment réglementé pour nos TPE à 280 euros le mégawattheure. Nous avons aussi une aide d'urgence Gaz et électricité mais aussi l'amortisseur qui va s'appliquer en plus des 280 euros le mégawattheure. Je veux vous dire que tout le coeur aujourd'hui de la mobilisation du gouvernement n'est pas tant sur l'ampleur 12 milliards d'euros sont à saisir l'argent est là, nous devons nous mobiliser pour dire à nos boulangers où se trouve le Z gouv Point FR sur la page d'accueil vous avez l'intégralité des coordonnées des conseillers départementaux qui sont là pour aider nos boulangers qui ont autre chose à faire que d'aller chercher les aides. Il faut qu'on se mobilise tous je connais l'engagement des sénateurs. Il y a le guichet il y a l'amortisseur. Il y a les 280 euros et il y a aussi des dispositifs d'étalement charges si nécessaire à votre disposition pour en reparler après je vous remercie. Merci la parole est maintenant Madame. Catherine Procaccia. Merci, monsieur le Président, bonjour, madame la Ministre. Ma question porte sur les nouvelles obligations pour les propriétaires de déclarer la situation de leurs biens immobiliers. La loi de finances pour 2020 oblige, d'ici le 30 juin, 34 millions de Français, a déclaré chacun de leurs locaux d'indiquer à quel titre ils les occupent l'identité des locataires et leur période d'occupation. Je m'étonne de l'absence de communication auprès des contribuables de cette nouvelle obligation qui en plus est sanctionné par une amende de 150 euros par local oublié. Sans compter que des caves et les parkings sont prévus comme des locales et apparaissent comme des biens indépendant. Sans compter que l'administration affecte automatiquement un pourcentage de parties communes qui ne sont pas en rapport avec les IM de la copropriété. Enfin le calcul des pièces ne correspond absolument aucune pratique habituelle puisque les salles de bain sont comptés comme des pièces les cuisines aussi et ça, quelle que soit la dimension pire en cas d'erreur et j'ai testé, il est impossible de corriger soi-même. Je souhaite donc savoir ce que vous avez prévu pour accompagner les Français dans ce processus qui est en cours d'heure otages semble-t-il ainsi que pour les personnes qui continuent à faire des déclarations papier.

sur un sujet que vous connaissez bien, je vous passe l'introduction puisque vous connaissez bien le sujet. Effectivement, les propriétaires, vous l'avez bien mentionné doivent indiquer à l'administration fiscale et ce avant le 1er juillet à quel titre ils occupent. Les locaux habitation principale ou secondaire et quand ne l'occupe pas eux-mêmes l'identité des occupants. En matière de communication parce que c'est le coeur de votre question. Plusieurs actions que je me permets de vous rappeler ont d'ores et déjà été réalisées et vont s'intensifier dans les prochains mois un message spécifique d'abord a été affiché en première page des avis de taxe foncière et de taxe sur les logements vacants à l'Automne 2022. Par ailleurs, un encart informant sur les nouvelles démarches et visible sur le site gérer mes biens immobiliers par ailleurs des actions de communication sont en cours auprès de la presse nationale locale télévision et radio et des campagnes d'information personnalisée ciblées. Vont être réalisées à partir du mois de février, via des mails et des courriers papiers je je comprends votre agacement. Au moins, même si on est un peu en retard, c'est en cours et c'est prévu pour février. Ces campagnes vont aussi s'accumuler avec la campagne de déclaration des revenus 2023. Qui va représenter également une étape importante pour communiquer auprès des usagers particuliers, comme pour toute réforme d'envergure, l'administration fiscale. Fera aussi preuve. De bienveillance. À l'endroit des propriétaires qui n'aurait pas été informé par ailleurs pour répondre à vos interrogations sur les informations restituer au sein du service géré mes biens immobiliers. Une dépendance en dehors des murs. ne vais pas, ça va être trop long, j'aurai pas le temps, ils m'ont fait un exemple très concret que je propose, madame la sénatrice Procaccia de vous transmettre après. À l'aune de désinformation sur le service géré mes biens immobiliers mais hein. Vous avez raison, il faut plus communiquer de ça arrive au mois de février. Espérons que ce soit suffisant. Votre question est fort légitime, je vous remercie. Madame Procaccia à 44 secondes. Merci. Alors effectivement la communication semble indispensable, la bienveillance aussi puisque c'est quand même un secteur qui était géré par l'administration et qui maintenant est reportée sur les particuliers. Madame la ministre, on est quand même très nombreux à ne pas aller régulièrement sur notre site des impôts hormis quand on a besoin de les payer, donc l'information est indispensable mais les le petit les calculs comme quoi. une salle de bain, même si elle fait un mètre carré demi est une pièce une entrée si elle fait 18 m2 n'est pas une pièce une cave est une pièce, c'est complètement aberrant et on ne peut pas corriger donc j'espère que. Ces éléments vont pouvoir être remis en cause et qu'on va s'quand même s'interroger un petit peu sur les ses modalités de déclaration. Ouais ben madame. Qu'est-ce qu'on sait encore. Là. Pour casser les pieds au monde. On est quand même champion du monde On est quand même champions du monde pour casser les pieds aux gens hein allez je dis ça je dis rien, mais alors moi moi je découvre. Et vous croyez que je vais sur le site. Comment vous dites, gère immobilier je sais pas quoi enfin qui y va là-dessus enfin franchement. Bof moi à part les payer. Bon enfin bref allez. La parole est à monsieur Didier Marie. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre je me fait aujourd'hui l'écho auprès de vous, de l'inquiétude du désarroi des boulangers de Seine qui sont confrontés à une explosion du montant de leur facture d'électricité. 60% des 3000 boulangeries que compte le département sont au tarif jaune et voient leur facture augmenter ceux qui renouvellent leur contrat connaissent des augmentations considérables qui ruine leurs marges. Les dispositifs d'aide que vous avez mis en oeuvre et que vous leur proposez n'apaise pas leur craintes pire suscite souvent la colère par le sentiment de ne pas être entendus. Le bouclier tarifaire limite certes à 15% la hausse du prix d'électricité en 2023 mais son bénéfice est subordonnée au nombre de salariés, moins de 10 et la puissance du compteur électrique. Or les boulangeries ont pour 80% d'entre elles des compteurs supérieurs à 36, qui veut qu'avait ah et il n'y sont donc pas éligibles. Les solutions alternatives, à savoir l'amortisseur électricité pour cette puissance de compteur la garantie que le prix du mégawattheure ne dépassera pas 280 euros et le fait de dépenser plus de 3% de leur CA en énergie ne répond pas aux difficultés ces dispositifs proposés aux boulangers ne sont pas à la hauteur alors qu'ils sont par ailleurs soumis à une envolée du prix des matières premières, plus 14% pour la farine, plus 30% pour le beurre plus 25% pour le sucre et caetera. Les conséquences de cette situation sont doubles, une augmentation du prix de la baguette à venir et toute la boulangerie qui frappera le pouvoir d'achat des ménages et contribuera à l'inflation et d'autre part des risques de suppressions d'emplois, certains l'ont déjà réalisé et la disparition d'un grand nombre de commerces. Sachant que le boulanger et dans bon nombre de nos communes rurales, le dernier à être ouvert. Madame la Ministre quelles dispositions nouvelles comptez-vous prendre pour sauver nos boulangeries et la baguette Patrimoine mondial de l'UNESCO. Merci madame la ministre. Merci monsieur le président, monsieur Didier Marie, j'ai l'honneur d'être la ministre des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, mais je ne suis pas à la ministre du commerce, de la peur. Je sais que c'est difficile. Vous faites bien de m'interroger et heureusement que la représentation nationale m'interroge mais ça fait plus de 6 mois que je sais que c'est compliqué et donc plus de plusieurs mois qu'on s'attelle à trouver des solutions. Je connais un peu et respecte beaucoup les socialistes pour savoir que contrairement à d'autres partis plus extrêmes. Vous ne vous voterez pas dans ce commerce de la peur et donc je pense comme je l'ai dit et je me suis permis de le dire, il y a juste un instant que notre devoir en tout cas je me permets de le partager n'est pas comme certains l'ont fait d'écrire à nos boulangers pour leur expliquer comment ils vont mourir. Mais d'écrire à nos boulangers en leur disant comment on peut s'en sortir. Je ne peux pas laisser dire. Que les mesures en tout cas que la prise en compte par le gouvernement de l'ampleur de la crise chez nos artisans boulangers. Elle est secondaire. Il y a 12 milliards d'euros à aller chercher au moment où je vous parle, on m'a parlé de l'Allemagne. On m'a parlé d'autres pays européens, il y a pas un pays en Europe qui a mis autant d'argent à disposition pour les entreprises. Les Allemands parlent de beaucoup d'argent au moment où on se parle, nous on a fait de choses hein, je vous ai entendu Monsieur le le sénateur Marie. Il dit on ne peut pas augmenter le prix de la baguette, ça va grever le pouvoir d'achat. Des consommateurs il y a pas un pays européen qui a fait ce qu'on a fait avec un bouclier qui est en fait un plan de relance de la consommation. Un bouclier tarifaire à 15% c'est 110 milliards d'euros pour soutenir le pouvoir d'achat des Français. Oui et nous assumons et la Confédération générale des boulangers d'ailleurs leur a dit, on peut augmenter de 3 5 %. Le prix de sa baguette, les consommateurs et des sur la facture d'énergie peuvent tout à fait supporter cette hausse l'État supporte l'immense majorité de la hausse des coûts de l'énergie à plus de 50%. Bercy l'a démontré, quasiment à 60% et aujourd'hui il y a une chose à faire et vous savez moi j'ai été plutôt plus entrepreneur que femme politique, alors des fois on me dit c'est compliqué. Allez sur impôts Point gouv Point FR sur la page d'accueil il y a rien à chercher il y a pas d'anglais. Monsieur le Président, sur la page d'accueil, on ne peut pas le louper. Vous avez l'amortisseur. Vous avez le guichet, vous avez le 06 les coordonnées directe des conseillers départementaux pour sortir de cette crise. Donc il y a des dispositifs d'aide notre mission. Ça doit être de les activer, aujourd'hui on est loin d'avoir décaissé. Moi je suis prêt à me battre et à me battre au-delà de tout. Mais une fois qu'on a décaissé c'est 12 milliards qui sont pour nos boulangers de grâce et des mois à leur dire qu'il faut signer cette petite attestation disant je suis une TPE j'une PME et juste à le renvoyer à son fournisseur pour bénéficier de ces aides avec ces aides on peut passer le moment difficile. On a des solutions, il faut que ces aides soient décaissés, on a un vrai problème de non recours mais 12 milliards d'euros. Ça n'est pas anodin. Et je peux vous garantir qu'on est là pour les décaisser je vous remercie. Merci, madame la Ministre 15 secondes monsieur Didier Marie. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre. Je crois que il y a un écart entre ce que vous dites et ce que ressentent et vive les boulangers de mon département comme vraisemblablement des autres départements. J'ai eu ce matin au téléphone le président des boulangers de Seine-Maritime qui m'a confirmé qu'un grand nombre de ses collègues étaient en grande difficulté et craignait de devoir licencier ou fermer leur boulangerie et donc le problème est réel et les aides que vous mentionnez ne sont pas suffisantes. non. Madame la Ministre pas de débat. Pas de débat. La parole maintenant Madame Jocelyne Guidez. Oui, merci Monsieur le le président Madame la Ministre, mes chers collègues, je souhaiterais attirer votre attention sur les difficultés administratives et financières rencontrées par nos soldats blessés français dans nos administrations pour un blessé du fait de son engagement militaire, il devrait exister une présomption de bonne foi nous devons alléger la charge de la preuve qui pèse sur l'individu. Nous devons même la neutraliser afin de mieux les accompagner, nous devons garantir à nos soldats et à leurs familles. Une prise en charge immédiate durable adapté et bienveillante pour reprendre un mot sans ambiguïté du président Emmanuel Macron lors de son discours du 13 juillet 2022 sur la politique de défense. Néanmoins nous constatons l'ampleur des difficultés de soda blessés, tous grades confondus dans leur parcours médico-administratifs ainsi que leur énorme déception de devoir parfois saisir le tribunal administratif afin de faire tout simplement valoir leurs droits lassés ils abandonnent souvent, n'oublions pas que cette action de simplification demandées par nos soldats ne serait qu'une simple expression de reconnaissance pour leurs sacrifices et leur engagement sans faille. La seule chose qui demande, c'est de pouvoir conserver leur dignité et être en mesure de subvenir dignement aux besoins de leur famille. Malgré leur handicap. N'oublions pas que toute blessure psychique physique ou neuropathique ou neuropathique a un impact significatif au quotidien. Madame la Ministre, malgré que vous soyez pas Ministre de excusez-moi des anciens combattants. Savez-vous quelle est la pensée malheureuse de nombreux soldats blessés, il vaut mieux être un soldat ayant été au sacrifice ultime qu'un soldat blessé puisque le décès de l'individu débloque toutes les instances. Ne serait-il pas temps de prendre en compte réellement de soda, blessés face à cette triste réalité. Je vous remercie. Merci madame la ministre. Merci madame la sénatrice et effectivement j'ai pas l'honneur d'être en charge des anciens combattants. Mais j'ai l'honneur. De connaître très bien le handicap et. Les drames de la vie et donc, votre question. D'abord me touche et je vais essayer d'y répondre avec le plus de précision possible en me faisant. La messagère si vous le souhaitez à l'endroit de la ministre en charge. Des anciens combattants de la prise en charge des blessés que vous mentionnez dépasse amplement le simple devoir moral. Et j'ai à coeur de de vous répondent nos militaires doivent pouvoir conduire de manière sereine. Les missions assignées sans avoir à redouter un 2ème parcours du du combattant et c'est bien pour ça. Que il est important de faire émerger la présomption de bonne foi en faisant oublier les processus administratifs désincarnées pour instaurer un accompagnement individualisé aussi bienveillant que possible la prise en charge déjà elle doit être simplifié. Elle doit être simplifié rapidement tout en développement, la dimension territoriale des dispositifs d'aide. Un nouveau plan d'action ministérielle d'accompagnement des blessés et des familles qui les placera au coeur de toutes les attentions et prêts à être déployés et s'attachera prioritairement à améliorer la prise en charge et le suivi dans le temps long. Des militaires blessés à réduire les démarches administratives qui pèsent sur eux. Il a mieux leur faire connaître les droits et dispositifs d'accompagnement et à améliorer les dispositifs de reconnaissance de réparation. Si les travaux entrepris ces dernières années, on contribue à réduire les délais de traitement des dossiers. Soyons clairs à madame la sénatrice. Il nous faut désormais simplifier encore beaucoup les procédures. Ça va passer notamment par l'élargissement des cas d'attribution automatique des droits mais aussi par la réduction du nombre de du nombre de démarches et par une meilleure accessibilité. Au au dispositif dont nos anciens combattants ont droit à travers des outils numériques et plus moderne. La ministre. Patricia Mirallès devrait présenter ce ce plan et surtout le déployer assez rapidement et à votre disposition si vous souhaitez que. C'est l'avantage de ces questions orales sans débat je lui en parle. En sortant de cet hémicycle, merci de votre question sur un sujet qui devrait tous nous mobiliser. Merci madame Guinness. 21 secondes. Merci monsieur le président, madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse. Il faut savoir quand même que la simplification. Ça fait au moins deux ans que je me bats là-dessus. Avant c'était madame Darrieussecq. Donc vous êtes en train de me dire que il y a un travail qui est fait actuellement. actuellement. Dommage que les parlementaires ne soient pas impliqués là là-dedans en tout cas c'est quelque chose qui m'aurait énormément intéressé et le fait que vous me dites que la réduction des démarches. Voilà, seront en tous les cas dans cette proposition me semble vraiment très important aujourd'hui. Merci. Merci la parole est à Madame Anne-Catherine Loisier. Merci monsieur le président, madame la ministre ma question porte sur les conséquences de la de libre-échange entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande sur la filière ovine. Le 30 juin 2022. La Commission européenne a acté la signature de cet acteur. Qui octroie donc un contrat. Un quota de 38.000 tonnes équivalent carcasse en plus des contingents déjà accordé historiquement à la Nouvelle Zélande concernant la viande congelée principalement ainsi la quasi-totalité de la viande ovine néo-zélandaise être importé sous l'appellation en frais à à des prix qui nous savons ne peuvent concurrencer nos éleveurs français soumis à des normes. Ces animaux sont en fait abattu en janvier pour être vendues en mars avril enfin pour pas qu'en France donc juste à la période où nos éleveurs ont prévu leur mise à bas sachant que s'ils n'arrivent pas à vendre leurs animaux mais elles sont obligés de les garder avec des surcoûts quant à leur entretien.

Les producteurs Madame la Ministre sont donc inquiets. De ses conséquences, des conséquences de cet accord qui vient dans une situation qui est déjà quand même tendu suite à l'accord avec

commerciaux sur des denrées pourtant disponible en France avec des pays situés de l'autre côté de la planète. Merci, madame la Ministre. Merci monsieur le président, madame la sénatrice Loisier. Je tiens d'abord à vous assurer que dans cette négociation commerciale. La France est particulièrement vigilante. S'agissant des intérêts de nos filières agricoles sensibles. L'ouverture du marché européen des viandes ovines était l'un des principaux intérêts de la Nouvelle Zélande et nous avons fermement défendu nos filières l'ouverture finalement accordé et de 38.000 tonnes, elle sera progressive, sur 7 ans et nous avons limité celle accordée aux viandes fraîches à 13.500 tonnes. Par ailleurs, la Nouvelle-Zélande est loin d'utiliser l'accès au marché européen dont elle dispose déjà par nos engagements à l'OMC le risque d'une augmentation des importations, avec ce nouvel accord et par conséquent relativement pour ne pas dire très faible. Ah fonctionnement normal de plus largement. Vous demander ce que le gouvernement fait pour rendre plus cohérentes les politiques européennes de durabilité et de commerce et je tenais à vous apporter quelques éléments de précision. Le rééquilibrage de la politique commerciale vers une meilleure intégration des enjeux de développement durable et très poussée par la France sous la présidence française de l'Union européenne. Le concept de mesures au mur miroir a d'ailleurs commencé à se généraliser. Il est important et vous le savez très bien, parce qu'il permet justement d'appliquer les normes de production européenne aux produits importés sur tous les flux commerciaux couverts ou non par désaccord il est juste. Essentiel ainsi. Nous saluons le fait que la commission a enfin présenté en décembre dernier, le projet d'actes permettant la mise en oeuvre de l'interdiction d'importer des viandes produites avec des antibiotiques comme facteur de croissance et nous nous félicitons aussi de l'accord récent sur la lutte contre la déforestation importée, enfin je voulais aussi souligné que l'accord avec la Nouvelle-Zélande et doté du chapitre commerce et développement durable plus ambitieux, négocié par l'Union européenne à date, il intègre l'accord de Paris comme élément absolument essentiel mais aussi la possibilité de sanctions commerciales en cas de violation substantielle de l'accord de Paris et des droits fondamentaux des travailleurs. Je vous remercie. Mais c'est Madame Loisier. Merci, madame la Ministre, les clauses miroirs son effet effectivement déterminante. Mais il n'en demeure pas moins aujourd'hui que nous éleveurs sont dans des situations catastrophiques et ne, n'arrive plus à, à vivre de leur production ce qui met en en en cause la souveraineté alimentaire de notre pays. Donc je pense que le sujet reste entier. Merci. Merci. C'est la parole est maintenant Monsieur Henri Cabanel. Merci, monsieur le Président. Madame la Ministre j'ai eu l'occasion d'échanger avec votre collègue de l'Éducation nationale au sujet d'une expérimentation que je propose dans mon département de l'Hérault. Il s'agit de créer des binômes d'élus parlementaires et élus locaux qui rencontreront périodiquement les jeunes de niveau élémentaire jusqu'au lycée. Même discours partout sans prosélytisme avec le seul filtre de l'information institutionnelle. L'éducation morale et civique ne remplit pas totalement ce rôle tant sur chien d'détermination s'est développé au fil des années, le tout dans une fourchette de temps très réduite. Le rapport d'information numéro 648 jeunesse et citoyenneté une culture à réinventer que j'ai déposée en juin 2022, s'est attaché à le démontrer. Des enquêtes auprès des jeunes également mon mon rapport propose d'organiser des une tradition d'élus de la République au sein des établissements scolaires dans un seul but de donner ces informations aux jeunes à partir d'un compte tenu établi par l'Éducation nationale. Car aujourd'hui de façon spontanée. Les élus interviennent dans les écoles, collèges ou lycées. Mais les contenus sont à leur propre initiative, il est primordial d'y mettre un cadre. Pourriez-vous Madame la Ministre valider cette expérimentation encadré par le rectorat, l'Association des maires de l'Hérault expérimentation qui sera réévaluée au bout d'une année scolaire. C'est madame la ministre. Merci monsieur le président. Monsieur le Sénateur Cabanel. La transmission, le respect des valeurs de la République sont au coeur de nos priorités de nos engagements. Dès l'école primaire tout au long de la scolarité, l'enseignement moral et civique permet aux élèves de mieux comprendre le bien-fondé de nos règles. Règles qui régissent nos comportements individuels mais aussi collectifs de mieux reconnaître le pluralisme des opinions. Des convictions, des modes de vie dans le cadre de cet enseignement mais aussi d'action éducative plus large des élus peuvent d'ores et déjà, oserais-je vous dire et je vais oser. Et heureusement. Et tant mieux intervenir auprès des enseignants pour apporter justement leur concours à cette transmission essentielle des valeurs de notre République. J'entends bien monsieur le sénateur, toute l'attention que vous portez au contenu. Et au bon déroulement de ces interventions qui impliquent des élus et accessoirement je la partage. Nul ne saurait en effet remettre en doute les bienfaits de ses interventions auprès des élèves. À condition qu'elle se déroule à l'abri de tout prosélytisme et dans le strict respect du principe de neutralité du service public de l'enseignement. C'est pourquoi, afin que ces interventions prennent tout leur sens, il est important comme c'est déjà le cas, qu'elles s'inscrivent. Dans le cadre du projet d'école ou d'établissement et qu'elles bénéficient, dans leur conception, mais aussi dans leur mise en oeuvre de l'appui des des équipes éducatives et pédagogiques des établissements dans lesquels elles ont lieu. Monsieur le sénateur, je vous remercie pour votre proposition qui concourt à l'éducation à la citoyenneté citoyenneté de nos élèves. Nous allons continuer à veiller comme vous, est-ce que ces interventions dans le cas de l'enseignement moral et civique s'inscrivent bien dans le cadre pédagogique adapté et surtout dans le cadre de la neutralité absolue du service public de l'enseignement, je vous remercie. Merci monsieur Cabanel. Merci madame la ministre je m'attendais à une telle riposte mais je vous l'ai expliqué dans dans la question. Un gros travail a été menée dans mon département avec la rectrice d'académie et. L'Association des maires de l'Hérault et j'ai justement pour éviter ce prosélytisme que j'ai, j'ai dénoncé ce que je dénonce moi aussi et que ça se fasse dans un cadre précis, porté par l'éducation nationale à travers le rectorat que je souhaite mener cette expérimentation et je sais, comme je vous l'ai dit que, effectivement, beaucoup d'élus le font mais là ça serait dans un cadre précis bien encadré et de façon à ce que toutes les écoles de notre département dans la durée des mandats des élus puissent en bénéficier. Voilà le but de cette expérimentation. Merci, cher collègue, la parole maintenant madame la présidente Annick Billon. Merci monsieur le président, madame la ministre ma question devait initialement porter sur la suppression de l'enseignement technologique, en classe de 6e ce sujet ayant été largement abordé la semaine dernière, je ne vais pas revenir dessus. En revanche je serai vigilante quant aux mesures qui émergeront des concertations qui sont en cours. Je souhaite donc vous interroger sur un autre sujet d'importance, les fermetures de classes et d'écoles en territoires ruraux. Alors que le gouvernement a présenté le soutien à la ruralité comme l'une de ses priorités. Plusieurs départements sont confrontés à des décisions unilatérales de fermetures de classes. Ces fermetures affectent de la carte scolaire du monde rural et pacte l'aménagement du territoire, envisagée par les élus et également forcément les projets d'investissement. Les propositions de l'État prévoit un abaissement du seuil de fermetures de classes ou d'établissements. Pour autant, il n'est pas acceptable que la baisse du nombre de postes inscrite dans la loi de finances pour 2023 puissent pénaliser en 1er lieu ces zones rurales dans lesquelles vous ne pouvez ignorer les difficultés liées à la mobilité cela fait d'ailleurs écho à l'engagement de l'État d'appliquer les mesures 73 74 de l'agenda rural, à savoir la prise en compte d'un indice d'éloignement et des prix spécificité des classes multi-âge aussi, quand et comment allez-vous appliquer ces mesures et ne plus imposer aux élus et aux familles des regroupements forcés dans des écoles des territoires ruraux. Je vous remercie, madame la ministre. Merci madame la ministre. Merci monsieur le président, madame la sénatrice Billon. Ça peut arriver, c'est assez rare mais. Nous pensions du, enfin du moins c'est les éléments dont je dispose que vous m'Roger. Sur l'enseignement en technologie. Et avec audace et. Heureusement que les parlementaires en non vous m'interrogez plutôt sur les fermetures de classes questions fort légitimes aussi mais dont il vous a pas échappé n'étant pas en charge du sujet, je n'ai pas une réponse satisfaisante à vous apporter du moins à mon sens, donc il y a 2 options, soit je vous fais une réponse. À côté de la plaque sur la technologie. Soit je suggère, comme je l'ai fait à 2 ou 3 reprises peut être de vous faire à apporter une réponse précise à la hauteur de la précision de votre question par le ministre de l'Éducation nationale. Ce que je peux m'engager à faire mais comme j'ai été longtemps enfin plus longtemps parlementaire que ministre j'aime pas répondre à côté de la plaque et je trouve que c'est pas. Hein c'est pas très respectueux. Donc si vous l'autorisez, je ferai une réponse écrite à une question orale mais je détestais compte j'étais au Parlement et que les ministres ils me répondaient bleu compte j'. Rouge, donc j'ai fait éviter de vous le faire. En revanche si vous acceptez de me transmettre votre question je vous garantis que je m'engage à vous apporter une réponse par le ministre de l'Éducation nationale. Rapidement, je vous remercie madame. La poésie ambition. Merci monsieur le président. Merci ma Madame la Ministre c'est tout à votre honneur. En réalité le le sujet est tellement récurrent dans les territoires que les questions se multiplient sur ce sujet il y a une demande de la part de l'AMRF 2ème question sur un moratoire. Il y avait eu un, un rapport d'un sénateur, il y a quelques années aussi Alain Durand qui disaient que oui on peut se dire qu'il y a eu une baisse de la démographie, mais on peut se dire aussi qu'on peut le le le l'objectif de son rapport. Donc peut-être que nous pourrions anticipée de et non pas d'avoir un couperet tous les ans qui tombe, je vous remercie, madame la ministre. Merci la parole est maintenant pour la dernière question madame Christine Herzog.

la suppression d'une classe de primaire de la commune de l'endroit en Moselle vient d'être décidé pour la rentrée 2023 sur décision du directeur académique des services de l'éducation nationale le d'Assen. Comme toute commune française, celle-ci a eu l'obligation d'ouvrir une école élémentaire publique selon l'article L 212 tiré de du code de l'éducation et d'en financer la construction, la maintenance et la mise aux normes, avec des remboursements à long terme. Ces articles fixe le seuil minima d'élèves obligatoire pour une, pour ouvrir une école à 15. Permettez-moi Madame la Ministre que je m'étonne de la fermeture d'une classe de 21 élèves. De plus, Les RPI sont marqués par des départs d'élèves sans dérogation. Ce qui est aussi le cas endroit qui a vu cinq enfants quitter ce dernier le manque de ses élèves jouent sous la décision des fermetures de classes. Une autre commune en Moselle Charlie Oradour matière pèse sur la fermeture d'une classe de maternelle, alors que la commune vient de viabiliser 93 terrains à bâtir. Or cette mesure de fermeture n'est pas sans conséquences. Sur les projets des familles et surtout sur les finances de la commune qui ont, qui voit son école fermer une classe qui n'est pas un signe de développement. Les phénomènes de fermetures de classes contribue à une désertification d'élèves dans les communes rurales Madame la Ministre lorsque les communes ou encore des engagements financiers des charges annuelles incompressible pour leurs écoles, comme c'est le cas de la commune de Land Charlie Oradour et etc et etc, la liste est longue. Pouvez vous suspendre les fermetures car ce sont 21 élèves par classe dont dispose l'école de la drogue et non pas 15. Selon l'article L 212 tiré de du code de l'éducation. Pouvez-vous différencier de seul d'élèves par classe, des zones urbaines et des zones rurales et ainsi faire des classes avec un maximum de 15 élèves en zone rurale et enfin pouvez-vous annulé les prises en charge les prises en charge des élèves 10 places déplacer et durcir les transferts d'accueil nos motivée je vous remercie. J'ai essayé de faire vite. Madame, mais si vous pouvez tout ça. N'hésitez surtout pas le dire. Si je pouvais tout ça tout en n'étant pas en charge de l'éducation nationale, ce serait. Ce serait presque même inquiétant. Monsieur le Président. Je je vous apporte madame la sénatrice Herzog quelques éléments de réponse. Sur ce sujet important. Déjà vous dire que le taux d'encadrement en Moselle a continué de s'améliorer en passant de 21 élèves par classe à la rentrée 2019. À moins de 20 élèves, 19, 8 élèves par classe à la rentrée 2022. Si on raisonne. À taux d'encadrement constant annuellement. À l'aune de ce que vous demandiez sur 15 élèves par classe en commune rurale. Si on arrive à des descendre de 2 élèves par classe par an, c'est un objectif que nous pourrions atteindre possiblement d'ici 3 4 ans s'agissant très particulièrement du département de la Moselle des 2 projets de fermeture en en d'école en zone rurale que vous mentionnez.

Alors moi j'ai Bourgas le trophée. Hé ben voilà donc je vous pouvez je suis nul voilà Guy Blin pardon mettent en place un regroupement pédagogique intercommunal avec une école à classe unique à 21 élèves répartis dans chacune des 2 communes ces de mer comme vous l'avez dit envisage de fermer leur école et scolariser leurs élèves dans la commune de benner strophes avec l'accord du maire. Le conseil municipal. De Galt trophée a acté la fermeture de l'école le 2 février dernier. Le conseil municipal de la commune de Guer. Ne s'est pas encore réuni sur la question. Pour l'instant sans les délibérations de tous les conseils municipaux c'est de retraits d'emplois ne sont pas actées par le directeur académique des services par le Dasen de l'éducation nationale, de la Moselle. Cette situation, madame la sénatrice Herzog fait l'objet d'un suivi très précis et attentif de l'inspectrice de la circonscription de Château-Salins. Dont dépendent les deux communes. Je suis cité et le ministère de l'Éducation nationale ne manquera pas de vous tenir informé. Je vous remercie. la séance sera reprise à 14h 30 pour le débat sur le thème l'État territorial entre mirage et réalité la séance, c'est sûr.